je voudrais excuser M. le Premier ministre, qui participe aux cérémonies commémoratives du soixante-quinzième anniversaire du débarquement allié du 6 juin 1944, comme il me l'a confirmé au téléphone ce matin. Je voudrais également excuser nos collègues sénateurs de Normandie, dont les présidents de commission MM. Philippe Bas, Hervé Maurey et Mme Catherine Morin-Desailly, ainsi qu'un certain nombre de sénateurs représentant les Français établis hors de France, qui ont l'honneur de représenter la Haute Assemblée lors de cette cérémonie. Il y a, en effet, exactement soixante-quinze ans, sur les plages de Normandie- territoire particulièrement cher à mon coeur -, des dunes de Varreville au port de Ouistreham, 136 000 hommes venus du ciel et d'une mer qui tentait de s'apaiser décidèrent, au fond, du sort de la guerre et, par-delà, de la liberté des hommes et des femmes et de l'avenir de la démocratie.

Ce jour-là, sur cette terre de Normandie, 3 500 sont tombés. Ces jeunes, souvent d'à peine 20 ans, dont beaucoup d'entre eux n'avaient jamais- ou si peu -entendu parler de la France, au milieu de cet enfer de feu et d'acier, n'ont pas hésité : ils ont avancé, avancé sur le sol de France, bravant les balles et les obus ils ont avancé, tombant les uns après les autres, pour abattre un régime diabolique ; ils ont avancé pour nous libérer. Parmi eux, figuraient les membres du bataillon Kieffer, dont le lieutenant de vaisseau Augustin Hubert, qui donna sa vie, parmi les premiers, à Ouistreham. Comment ne pas avoir une pensée pour nos marins tombés voilà quelques jours en Afrique, héritiers

Ce débarquement est à jamais inscrit dans nos esprits par tant de souvenirs, tant de livres et tant d'images. C'est sur ces plages qu'une certaine manière de vivre, de croire et d'espérer l'a emporté sur le seul, le véritable ennemi : le nazisme. Aujourd'hui, dans le respect de l'histoire et des souffrances éprouvées- je veux aussi avoir une pensée, pour des raisons que certains comprendront, pour les populations civiles si durement éprouvées dans ces nuits du 5, du 6 et du 7 juin, en cette terre de Normandie -, l'heure est d'abord au recueillement et au souvenir. Elle est aussi à ce présent que nous avons choisi de construire en commun, dans la diversité de notre démocratie. Au fond, l'idée européenne, les projets qui l'incarnent sont sont peut-être nés sur les plages de Normandie. Oui, ils sont nés sur les plages de Normandie, avec la liberté et la démocratie restaurées, avec le sentiment unanime que ces guerres fratricides qui ont enflammé le monde étaient la négation de l'Europe, de ses valeurs et de sa culture, avec le sentiment que tant de souffrances et de destructions ne pouvaient avoir été endurées en vain, avec le sentiment que nous devions à ces morts, dont beaucoup reposent aujourd'hui en Normandie, de donner un sens à leur sacrifice en nous engageant résolument dans la seule voie qui assure la paix

! Par lettre en date du 6 juin 2019, le Premier ministre, M. Édouard Philippe, m'a informé que M. François de Rugy, ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, présentera, mercredi 12 juin, le texte de la déclaration de politique générale qu'il prononcera au même moment devant l'Assemblée nationale. Par ailleurs, le Premier ministre demandera au Sénat l'approbation de cette déclaration en application de l'article 49, alinéa 4, de la Constitution. Acte Je réunirai la conférence des présidents mardi prochain, afin de modifier en conséquence

Cette dynamique s'est aussi traduite par des projets d'investissement étrangers. Avec 1 027 projets d'investissement sur son sol, dont 339 dans l'industrie, la France est le deuxième pays le plus attractif d'Europe, après le Royaume-Uni, mais devant l'Allemagne. Nous nous réjouissons de cette tendance positive, mais nous restons prudents quant à l'avenir de l'industrie française. La France et l'Allemagne doivent publier prochainement un document de politique industrielle européenne, comprenant notamment une proposition de réforme des règles de la concurrence.

vite proposée, mais aussi vite retirée. Sans fusion, et encore plus en froid avec son partenaire Nissan, Renault n'est-il pas aujourd'hui dans une situation plus fragile qu'avant ?

D'autres acteurs sont dans une situation préoccupante : Ascoval est en sursis. Le choix et l'analyse du repreneur étaient-ils pertinents ? Le premier n'a pas permis d'aboutir et le second est lui-même en difficulté. Je voudrais saluer ici le courage des salariés, qui restent dignes dans cette épreuve. Les différentes interventions de l'État sur Whirlpool, sur Alstom, sur General Electric et sur Ford n'ont pas permis d'empêcher les licenciements.

J'avais fixé, depuis le premier jour, quatre conditions au succès de cette opération : qu'elle se fasse dans le cadre de l'alliance entre Renault et Nissan, que l'emploi industriel soit protégé, que la gouvernance soit garantie et que la future entité participe au projet de batteries électriques que nous avons lancé avec l'Allemagne. Certaines de ces garanties étaient remplies ; l'une ne l'était pas, celle du respect de l'alliance entre Renault et Nissan. Nissan n'étant pas prêt à voter au conseil d'administration de Renault en faveur de cette fusion, nous avons demandé quelques jours supplémentaires pour discuter avec la partie japonaise et pouvoir lancer ce projet de fusion dans les meilleures conditions possible. Fiat a fait le choix de retirer son offre. Nous considérons qu'il était indispensable que ce projet se réalise dans le cadre d'une alliance entre Renault et Nissan, laquelle, depuis vingt ans, a apporté technologie, emploi et sécurité financière à Renault. Quel est maintenant l'avenir de Renault ? Tout d'abord, je tiens à redire qu'il s'agit d'une entreprise solide, performante. Ensuite, il faut consolider l'alliance entre Renault et Nissan. La direction va s'y employer. Je pars moi-même pour Tokyo dans quelques instants ; je vais aussi m'y employer avec mon homologue japonais. Enfin, nous restons ouverts à toute perspective de consolidation industrielle, mais, une fois encore, dans la sérénité, sans précipitation, pour garantir les intérêts industriels de Renault et de la nation française.

Le 12 mai dernier, les élections provinciales de Nouvelle-Calédonie ont permis de renouveler les assemblées de province et le Congrès. La famille politique à laquelle j'appartiens a largement remporté ce scrutin : avec avec 41 % des voix dans la province sud, elle y occupe désormais vingt des quarante sièges à pourvoir. Nous avons également obtenu trois sièges dans la province nord, à majorité indépendantiste. Ce scrutin vient confirmer les résultats du référendum du 4 novembre dernier, à l'occasion duquel le «

mais aussi à la France, à nous qui sommes dans cet hémicycle et qui incarnons la représentation nationale. Malgré ces résultats, la Nouvelle-Calédonie se retrouve aujourd'hui dans une situation totalement absurde. Par un jeu d'alliances,

Pour la majorité des Calédoniens, cette situation est incompréhensible, voire intolérable. Cette majorité a le sentiment que les résultats du référendum et des élections du 12 mai lui ont été confisqués et que son choix d'un avenir dans la France est ignoré. Cette majorité a même l'impression qu'on l'emmène subrepticement là où elle ne veut pas aller. Monsieur le Premier ministre, pour clarifier cette situation et avant qu'elle ne dégénère, les élus

Aujourd'hui, les présidents et vice-présidents des provinces ont été élus, ainsi que le président et les responsables des instances du Congrès de Nouvelle-Calédonie. Ce dernier vient d'ailleurs de se prononcer sur le nombre de membres du gouvernement de Nouvelle-Calédonie.

Madame la secrétaire d'État, au moment où le Sénat se penche sur l'avenir de la filière sidérurgique à travers une mission d'information qui rendra ses conclusions mi-juillet, je souhaite vous interpeller sur la situation de l'aciérie Ascoval de Saint-Saulve, dont le savoir-faire est reconnu par tous. Comme vous le savez, les salariés d'Ascoval ont rencontré, en début de semaine, le repreneur, M. Marc Meyohas, président de Greybull. Je tiens, à mon tour, à saluer le courage et l'exemplarité du comportement des salariés, qui sont aujourd'hui fatigués et lassés de toutes ces incertitudes. Le repreneur Greybull Capital est également le propriétaire de British Steel, groupe industriel britannique placé en redressement judiciaire.

Tout en saluant le travail considérable mené par le ministère, je souhaite vous interroger sur la stratégie que vous avez choisi d'adopter pour permettre au gouvernement français d'accompagner cette filière. Avez-vous des échanges avec vos homologues britanniques pour anticiper la reprise de cette unité de British Steel par un repreneur qui pourrait être- ce qui serait le meilleur scénario industriel -Ascoval et son repreneur ? Quels moyens l'État mobilise-t-il pour assurer un avenir à cette filière ?

ces hauts fourneaux vont perdre l'accès au marché européen et ne bénéficieront plus des mesures de protection qui avaient été mises en place pour protéger l'acier de l'Union européenne contre des sur-exportations de certains pays, notamment la Chine.

c'est un signe de confiance. Pour répondre à votre question, oui, nous accompagnons Ascoval, nous lui donnons toutes les garanties et lui renouvelons notre soutien dans cette démarche

Je partage bien entendu le constat général sur la situation budgétaire de notre pays : nous avons besoin de réduire les dépenses. Il y va indéniablement de notre crédibilité vis-à-vis des investisseurs étrangers, qui, selon les derniers chiffres, réinvestissent fortement grâce à la politique menée par le Gouvernement depuis deux ans.

Vous le disiez vous-même, les associations représentent un trésor, un trésor qu'il nous faut préserver. À l'heure où l'on évoque des ajustements quant à la fiscalité du mécénat et du don, il faut agir avec mesure et précision. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en modifiant la fiscalité, même légèrement, on peut provoquer des changements de comportements chez nos concitoyens qui impactent radicalement nos trésors associatifs. nos trésors associatifs. À l'heure où certains s'inquiètent de la situation financière de nos associations et de la baisse des dons enregistrés ces deux dernières années, pouvez-vous nous dire ce que vous comptez faire pour répondre à ces inquiétudes légitimes ? La parole

Le 1 juin, les prix de l'électricité ont augmenté de près de 6 %. Cette augmentation considérable devrait encore être amplifiée en août prochain. Pour un foyer qui se chauffe à l'électricité et dépense annuellement en moyenne 1 500 euros, cette hausse représentera un surcoût de près de 90 euros. Vous avez annoncé que la formule de fixation du prix de l'électricité serait revue à l'occasion de l'examen du projet de loi sur l'énergie, qui doit intervenir dans les prochaines semaines. Mais derrière la révision d'une formule technique, il y a d'abord une volonté politique. Elle consiste à donner des instructions pour aller dans un sens ou dans un autre afin de protéger certains plutôt que d'autres. Plusieurs associations de consommateurs ont mis en évidence que cette hausse est deux fois supérieure à l'augmentation des coûts d'EDF, qui s'élève à 3 %, le surplus de hausse servant à favoriser la bonne santé des concurrents d'EDF. L'Autorité de la concurrence avait d'ailleurs rendu un avis défavorable à la proposition de la Commission de régulation de l'énergie en soulignant les fragilités juridiques. Lors de l'examen du projet de loi que j'évoquais, nous discuterons pour savoir ce qui doit justifier le coût de l'électricité. Nous trancherons sur ce qui doit être consacré à la transition énergétique, laquelle suscite beaucoup d'attentes chez nos concitoyens. Nous discuterons aussi du coût du nucléaire, sachant que l'entretien et la sécurité des centrales ne sont pas négociables. Alors que, dans quelques jours, nous débattrons d'une proposition de loi sur la question de la précarité énergétique, je crois pouvoir dire que nous serons attentifs à ce que ce ne soient pas que les plus modestes qui paient. Or ceux-ci sont particulièrement exposés. En effet, leurs logements sont mal isolés isolés et les taxes qui pèsent pour un tiers sur le prix de l'électricité sont également soumises à la TVA, impôt particulièrement injuste, car il frappe sans distinction toutes les classes de la société.

Dans le cadre de sa réforme constitutionnelle, le Président de la République souhaite inscrire dans la Constitution la préservation de l'environnement. Nous avons entendu la préoccupation de votre majorité vis-à-vis du réchauffement climatique,

Allez-vous annoncer un plan de réinvestissement qui permette de relancer le fret ferroviaire en France, durement impacté depuis son ouverture à la concurrence en 2006 ?

qui transporte aujourd'hui ces fruits et légumes en provenance du sud de la France depuis la plateforme de Perpignan jusqu'à Rungis, les plateformes de Rungis et de Perpignan et les clients de ce

le sénateur, nous sommes engagés dans une politique de développement du transport ferroviaire. Nous n'avons jamais autant investi dans le rail en France qu'en cette période.

Mme la sénatrice Létard le disait tout à l'heure à propos d'Ascoval : les commandes de rails pour régénérer les voies ont été multipliées par deux. C'est du concret ! Cela signifie qu'on rénove deux fois plus de rails aujourd'hui qu'on ne le faisait auparavant.

de marchandises utilisent davantage le train et moins le camion. En l'occurrence, pour ce qui est de Rungis, la SNCF s'est engagée à poursuivre le service ... Il faut conclure ! ... jusqu'à la fin de l'année, aux mêmes conditions, et à faire des propositions concrètes pour poursuivre le service les années suivantes.

les locomotives, on les a ! Dès demain, on peut louer des wagons neufs réfrigérés pour acheminer les 1 400 tonnes de fruits et légumes au MIN de Rungis. La SNCF est prête

Demain va s'ouvrir la Coupe du monde féminine de football. L'engouement populaire est fort et les attentes sont importantes pour notre équipe nationale. En 2024, ce sont les jeux Olympiques et Paralympiques que Paris va accueillir. Des événements qui consacrent l'élite du sport tout en suscitant une attente collective énorme.

provoque une crise dont le dénouement est impératif pour regagner la confiance du monde sportif. Tout cela sans oublier la baisse significative du CNDS. Dans nos territoires, l'inquiétude est palpable. Sous couvert de donner une plus grande autonomie aux fédérations et aux collectivités, cette orientation ne cache-t-elle pas une forme de désengagement de l'État ? Comment pourra-t-on former la future génération de sportives et sportifs sans l'aide publique de l'État ? Devra-t-on passer par des structures payantes, privées, à but lucratif, qui feront la part belle aux disciplines en vogue, oubliant les activités moins médiatisées ? Votre projet semble casser notre modèle national. N'est-il pas en train de briser toute la dynamique sportive, de nous faire courir le risque d'un déclassement dans les prochaines années ? Êtes-vous certaine de favoriser l'excellence et la renommée du sport à la française ? Nous aurions pu lever ces interrogations si un vrai débat parlementaire avait eu lieu. Madame la ministre, je vais vous poser quatre questions : où en est le programme Sport et société ? Où en est la mise en oeuvre de l'institut du sport pour tous ? Comment l'Agence nationale du sport va-t-elle se décliner dans nos territoires ? Pourquoi maintenir votre position sur le détachement d'office des conseillers techniques et sportifs ?

les collectivités locales n'existaient pas et le monde économique ne s'intéressait pas au sport. Depuis, le monde a changé, les attentes des Français aussi. Répondez aux questions, madame ! Aujourd'hui, une majorité de Français fait du sport en dehors d'un club. Surtout, un Français sur deux ne pratique aucune activité physique. Il était devenu impératif de requestionner notre modèle. C'est parce que les acteurs du monde du sport se sont démultipliés que l'Agence nationale du sport a été créée. Avec ce nouvel opérateur, l'État garde la main, mais il la tend effet, le sport, c'est, outre le haut niveau, le moyen d'être en bonne santé, de s'épanouir, d'éduquer ou de réparer. Cette agence marchera bien sur ses deux jambes : la haute performance et le développement du sport pour tous. madame ! Elle aura pour mission de piloter le déploiement des politiques sportives en concertation avec tous les acteurs et au plus près des territoires. L'État doit être plus agile et capable de s'adapter aux besoins de chaque Français. Et les conseillers techniques ? La création de l'Agence traduit aussi une nouvelle ambition, un État stratège et partenaire. Elle augmente la capacité d'action du ministère des sports, qui va assurer pleinement ses missions de sécurité des pratiquants, de respect des règles et d'éthique, de l'intégrité, de la formation, de l'élaboration de politiques interministérielles. Le ministère des sports conserve son rôle central dans l'élaboration, le pilotage et la mise en oeuvre des politiques publiques. J'entends dire, comme vous l'avez dit, monsieur le sénateur, que, depuis mon arrivée, le ministère des sports serait affaibli. Oui ! Permettez-moi, mesdames, messieurs les sénateurs, de le répéter devant vous, je suis fière de l'action d'un Gouvernement qui fait le choix fort de développer des politiques sportives ambitieuses et qui le traduit par un ministère des sports de plein exercice, ... Votre budget, madame ! ... chose qui n'est pas arrivée depuis un certain temps ; ... Il faut qui permettra de vous présenter une exécution budgétaire 2018 à son plus haut niveau depuis dix ans ; de l'action d'un Gouvernement ... Il faut conclure ! ... engagé derrière Paris 2024 pour en faire un grand événement populaire ; des politiques sportives et un ministère des sports ...

d'aménagement du territoire. Lors de la restitution du grand débat, M. le Président de la République a déclaré : « Les Français ont confiance dans leurs élus locaux et ce nouvel acte de décentralisation doit porter sur des politiques de la vie quotidienne », dont le transport, « pour garantir des décisions prises au plus près du terrain. » Il avait bien compris que le détonateur de la crise des « gilets jaunes » avait été le prix du carburant. À l'occasion de la loi Mobilités, un tir en règle s'est déclenché contre les petites lignes aériennes intérieures à travers des amendements visant à demander une nouvelle contribution au décollage et la suppression de la quasi-totalité des lignes. Vous n'ignorez pas que ces petites lignes ont un rôle essentiel de désenclavement pour ces territoires éloignés. Je pourrais citer Aurillac, Le Puy, Biarritz, Clermont-Ferrand et d'autres. J'affirme que, contrairement aux dires des auteurs de ces amendements, ces lignes sont empruntées non par des privilégiés mais en majorité par des acteurs essentiels de l'économie locale. Madame la ministre, quelle est la position du Gouvernement face à ces attaques contre des territoires enclavés et que proposez-vous ? Le Gouvernement est-il prêt à s'engager à renoncer à toute taxation supplémentaire ou interdiction qui pénaliserait une fois de plus l'aménagement du territoire ?

remercie, monsieur le ministre d'État, mes inquiétudes sont un peu levées, mais pas tout à fait. Pas d'autoroute, pas de TGV, parfois pas même de train- si vous avez la chance d'être à deux ou trois heures d'une gare de TGV, celui-ci est régulièrement en retard et souvent complet

des Français sont attachés à la liberté de choisir entre allopathie et homéopathie. Trois quarts des Français interrogés pensent que l'homéopathie a prouvé son efficacité et sont favorables au maintien de son remboursement.

Par ailleurs, l'homéopathie est un recours indéniable auprès des enfants et des femmes enceintes. Elle est aujourd'hui utilisée quotidiennement comme soin de support aux traitements anticancéreux. Ne plus la rembourser engendrerait une surconsommation de médicaments allopathiques et une augmentation de la charge financière supportée par notre système de santé. Enfin, économiquement parlant,

ont tous fait le choix de l'Hexagone pour la production de leurs médicaments : ils emploient plus de 3 200 personnes réparties sur l'ensemble du territoire national. Une telle décision aurait donc également des conséquences sociales particulièrement fâcheuses. Votre question ? J'y viens, monsieur le président. pouvez-vous nous indiquer si vous allez, ou non, dérembourser ces remèdes médicaux naturels et peu onéreux qui permettent de réduire la consommation allopathique ?

Depuis les années soixante, l'homéopathie bénéficie d'un statut et d'un régime dérogatoires. Il était important de mettre fin à ce débat en mobilisant une expertise scientifique et indépendante qui se baserait sur une analyse de la totalité de la littérature. C'est pour cette raison que Mme la ministre a saisi la Haute Autorité de santé en août 2018.

évidemment à ce sujet. Nous comprenons celles et ceux qui s'inquiètent, au sein des territoires, des risques que ce déremboursement pourrait avoir sur l'emploi et sur l'économie locale. Les laboratoires pharmaceutiques

Vous ne pouvez ignorer ni cette pratique ancestrale ni ces femmes et ces hommes qui, chaque jour, font vivre une économie locale prônant l'excellence, entretiennent nos paysages, garantissent le maintien des populations montagnardes et valorisent l'économie touristique. Ces éleveurs sont à bout de forces. Ils ne supportent plus de vivre sous une perpétuelle menace de prédation, à mesure que l'ours ou le loup se rapprochent des villages, que ce soit dans les Pyrénées ou dans les autres territoires de montagne. Ils n'en peuvent plus qu'on réponde aux attaques que subissent leurs bêtes par une indemnisation qui sonne comme un aveu d'échec. Ils n'ont que faire des mesures de protection, qui sont inefficaces face aux prédateurs dont le comportement est inquiétant. L'une des meilleures garanties contre la prédation est la présence humaine. Allons-nous, alors, condamner nos éleveurs à travailler dans des conditions archaïques, à 2 000 mètres d'altitude, nuit et jour, pour protéger eux-mêmes leurs troupeaux ? Face à la crise des vocations qui se profile, l'heure n'est plus aux mesures de prévention : il faut agir ! Un seul ours a récemment perpétré trois attaques en moins de cinq jours, à quelques centaines de mètres des habitations. Il a été présenté par les autorités comme anormalement prédateur. Aussi, monsieur le ministre d'État, à quand une étude mesurant l'impact économique, sanitaire et social de ces réintroductions ? Jusqu'où êtes-vous prêt à aller dans la mise en place des protocoles « ours à problème » ? Plus globalement, quand allez-vous entendre ces éleveurs et tenter de comprendre leur détresse ? La parole

Nous avons même procédé à la réintroduction de deux ourses slovènes, à l'automne dernier, dans les Pyrénées-Atlantiques, car nous voulons préserver l'ours des Pyrénées. Il n'y a qu'une dizaine qu'une dizaine d'ours dans l'ensemble du massif pyrénéen, ce qui rend de toute façon sa préservation fragile. Je vous le dis clairement, comme je l'ai énoncé aux éleveurs et aux élus locaux que j'ai rencontrés : nous ne mènerons pas une politique d'éradication de l'ours dans les Pyrénées. Nous sommes en revanche au rendez-vous pour

Maryse Carrère, pour la réplique. Si les éleveurs boycottent aujourd'hui la réunion de Toulouse, il y a bien une raison : ils ne croient plus en ces mesures de prévention

Les 436 missions locales constituent le service public territorial de l'insertion et de l'accompagnement des jeunes par excellence. Elles accompagnent 1,3 million de jeunes, dont 584 000 accèdent à l'emploi, 40 000 à un contrat en alternance, 186 000 à une formation professionnelle et 223 000 à une immersion professionnelle. L'action des réseaux des missions locales se trouve déstabilisée depuis plusieurs mois : l'accompagnement de centaines de milliers de jeunes Les responsables des missions locales de mon territoire du Pas-de-Calais m'ont fait part de leurs inquiétudes, relayées également par les élus locaux. Ils craignent une menace politique de fusion ou de contrôle des missions locales par Pôle emploi, ou encore une reprise des missions par des opérateurs du

Nos questionnements face au devenir des missions locales se nourrissent, malheureusement, de vos orientations politiques néfastes : la politique de l'emploi se trouve affaiblie par la réduction drastique des emplois aidés, qui touche les plus fragiles, mais aussi par la baisse des crédits et des effectifs alloués à Pôle emploi, décidée sous le prétexte d'une amélioration des chiffres de l'emploi, amélioration malheureusement très peu visible et très peu ressentie par les plus exclus de nos concitoyens. Ce lundi 3 juin, les 72 missions locales franciliennes ont organisé une journée morte pour dénoncer la baisse de leur financement pour 2019, baisse qui menace 70 emplois et, surtout, réduit les capacités d'accompagnement pour 10 000 jeunes. Ma question est simple et directe : quand allez-vous cesser de détruire méthodiquement tous les outils de la politique de l'emploi permettant aux plus fragiles de sortir de la spirale du chômage ?

je vous prie d'excuser Muriel Pénicaud, qui est retenue par le G7 social qui se tient, pendant deux jours, à son ministère. Je voudrais vous remercier de votre question : je partage vos déclarations sur le rôle important des missions locales, qui constituent un maillon essentiel du service public de l'emploi. Elles permettent de repérer, d'accueillir, d'orienter et d'accompagner les jeunes en difficulté. À ce titre, Mme la ministre du travail a souhaité que l'effort financier de l'État en faveur des missions locales soit préservé en 2019, malgré la contrainte budgétaire que nous connaissons. La répartition de ces crédits dépend des services du ministère du travail en régions, selon des critères qui prennent en compte les résultats des missions locales,

le précédent système et, d'ores et déjà, de résoudre les difficultés observées. Madame la sénatrice, nous partageons le même objectif, l'emploi des jeunes. Pour mener cette bataille, il faut que les missions locales continuent et amplifient leurs actions auprès des jeunes,

L'aménagement numérique du territoire fait partie des engagements du Président de la République. S'il faut bien reconnaître au Gouvernement une volonté de mettre en oeuvre des solutions efficaces sur le mobile, notamment par le biais du, en revanche, concernant les lignes fixes, les interventions semblent pour le moins incohérentes et leur efficacité très incertaine relever d'un pari hasardeux que de choix mûrement réfléchis. L'accélération promise se traduit en effet, en dépit d'une habile communication, par la relégation du 100 % FTTH pour tous vers un horizon de date qui recule au fur et à mesure que l'on s'en approche. J'en veux notamment pour preuve l'apparition de cette date de 2022 dans les nouvelles versions des conventions des zones dites AMII, alors que, jusqu'à présent, les opérateurs privés devaient inscrire leurs intentions dans un calendrier arrêté au 31 décembre 2020. Certes, des engagements valent mieux que des intentions, mais c'est ce que verront les habitants qui nous intéresse au premier chef. Quant aux résultats de l'accélération dans les zones dites AMEL, ils brillent par leur absence. vous avez présenté à Cahors, le 14 décembre 2017, ce nouveau dispositif temporaire comme devant se terminer à la fin de mai 2018. Or, retard après retard, il aura fallu dix-huit mois au Gouvernement pour accepter les trois premiers dossiers. Plutôt que d'accélération, il convient de parler de précipitation ! Dans le même temps, les réseaux d'initiative publique ont fortement accéléré leur déploiement, renégocié favorablement leurs contrats de DSP existants, ou en ont attribué de nouveaux, toujours plus favorables et économes en argent public. Il convient de clore les aventures hasardeuses de l'État et de rouvrir le guichet de financement du plan France très haut débit, afin de relancer la seule mécanique qui fonctionne à présent et qui offre toutes les garanties à l'État comme aux collectivités pour atteindre le 100 % FTTH : les réseaux d'initiative publique. Vous l'avez vous-même reconnu récemment par écrit, en indiquant que la fermeture du guichet était nécessaire pour que les AMEL aient une petite chance de succès. Cette chance est passée ! Votre question ! Le bilan est décevant, certes, mais l'important est maintenant de tourner la page, et de la tourner très vite. Monsieur le Premier ministre, rouvrez immédiatement le plan France très haut débit. Il est urgent de remettre de la cohérence, de la pérennité et de la visibilité dans l'aménagement numérique, pour le dynamisme et l'attractivité de notre territoire, et de cesser de jouer aux apprentis sorciers. Terminez ! Il y va de la crédibilité du Gouvernement en la matière

qui offre à tous les Français un accès au très haut débit et à des services mobiles de qualité. Depuis deux ans, le Gouvernement s'est donné les moyens de mettre en oeuvre, en pleine collaboration avec l'ensemble des acteurs, dont les élus locaux, les objectifs ambitieux définis au niveau national. Nous constatons que nos efforts sont payants : l'accélération des déploiements est une réalité, dans les zones urbaines comme dans les zones rurales. Chaque jour ouvré, 13 000 lignes en fibre optique sont construites. Cela représente 3,2 millions de lignes FTTH en 2018. Les chiffres du premier trimestre de 2019, qui seront annoncés demain, marquent une très forte accélération. Les collectivités territoriales ont fortement contribué à cette performance, en construisant près de 750 000 lignes de fibre optique en 2018, ce qui constitue un record pour les réseaux d'initiative publique. Pour l'État, ce programme représente un effort financier de 3,3 milliards d'euros. Dans l'Ain,

qu'il fallait, avant toute décision, vérifier dans quelle mesure les acteurs privés que vous avez évoqués étaient prêts à financer à leurs frais le reste des prises non financées. On parle là de 3 à 4 millions de prises, sur un total de 34 millions. Vous n'ignorez pas que j'ai fixé au 15 juin nous faire part de toutes leurs intentions d'investissement ; c'est une date finale, comme vous l'avez rappelé vous-même. À partir de là, nous ferons un diagnostic précis,

à nos côtés, pour un meilleur aménagement numérique de notre territoire.

Pourtant, comme l'Italie de Salvini, la France ne respecte pas ses engagements européens, car elle ne réduit pas son déficit structurel. Comme l'Italie de Salvini, la France choisit de baisser les impôts, aggravant ainsi les déficits. Comme l'Italie de Salvini, la France a un haut niveau de chômage réel et structurel : les mêmes causes produisent les mêmes effets. Comme l'Italie de Salvini, le Gouvernement choisit la dette, au risque de faire porter une menace je cite sur ce point le FMI. Alors, madame la secrétaire d'État, pensez-vous avoir raison, seuls contre toutes les institutions dont nous sommes membres ? Pensez-vous que la bonne politique économique soit celle de M. Salvini ?

était de ce point de vue en pole position dans la zone euro. La mission qu'a conduite le FMI du 20 mai au 3 juin a noté que la refonte du code du travail et celle de la fiscalité du capital sont des réformes importantes, qui contribuent à la résilience de l'économie. a précisé que les mesures en faveur du pouvoir d'achat ont un coût budgétaire. Il va donc falloir réduire les dépenses publiques pour appuyer les choix sociaux faits cette année. Je vous rappelle que nous assumons parfaitement ces choix sociaux

en amélioration par rapport à la prévision. S'il est vrai qu'il sera cette année supérieur à 3 %, c'est que nous devrons absorber des décisions liées au CICE qui ont été prises sous la mandature précédente. C'est factuel ; je tiens

Alors, oui, il faut admettre que la situation économique de la France progresse, que le chômage a baissé de manière significative, puisqu'il est à son plus bas depuis dix ans, et que- plus intéressant encore -le taux d'emploi est à son plus haut depuis quarante ans. La précarité aussi ! Pour ma part, je crois que cette politique économique réussit, et je suis fière de faire partie de ce gouvernement

Alors, le nouveau monde sera-t-il, en vérité, celui que vous menacez de préparer après une nouvelle crise économique ? Voulez-vous, par ce genre de politique, que nous nous réveillions italiens ?

Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée,

tout ce qui relève de l'organisation territoriale des établissements de santé, en l'espèce des hôpitaux de proximité. Alors que notre pays est touché par de réelles fractures sociales et territoriales, le Gouvernement ne doit pas être autorisé à faire l'impasse sur le débat parlementaire et à décider seul sur des sujets aussi majeurs que ceux de la carte hospitalière ou des modalités de gouvernance des établissements ayant obtenu le label « hôpital de proximité ». Nul ne peut ignorer la tendance comptable et centralisatrice qui a permis ces dernières années de réduire l'activité de certains hôpitaux faute de moyens, puis, à terme, d'organiser leurs fermetures par manque d'activité. De nouvelles fermetures de maternités, de services d'urgences chirurgicales et, plus largement, d'établissements sont à craindre. En l'état actuel du texte, trop imprécis, il n'est pas envisageable que le Gouvernement sursoie à débattre avec les parlementaires, représentants du peuple, de tels enjeux de santé publique et d'aménagement du territoire.

À défaut de débats sur la détermination des critères, nous demandons que les associations d'élus locaux et les principales organisations syndicales de la santé soient au moins consultées dans la définition des modalités selon lesquelles la liste des établissements de santé de proximité sera établie.

Les élus locaux, pourtant directement concernés et impliqués dans ce qui peut concerner les établissements de santé, notamment au regard de la lutte contre les déserts médicaux, ont perdu, avec la suppression des conseils d'administration des hôpitaux, toute responsabilité dans l'organisation stratégique de ces derniers. Ils ne demandent pas à avoir une voix prédominante sur les décisions purement médicales. Il est cependant inconcevable de ne pas reconnaître que les décisions relevant de l'accès aux soins ont aussi systématiquement un impact sur les territoires en termes de transports, de services, d'emploi, d'installation des ménages ... C'est pourquoi la question de la gouvernance des hôpitaux de proximité devra être traitée à l'occasion de la rédaction des ordonnances annoncées, qui devront nécessairement être élaborées en concertation avec les associations

est favorable. Tout va bien ! Continuons comme ça ! Les personnels sont en lutte et se bagarrent dans la rue pour obtenir une rencontre avec Mme la ministre, qui les a peut-être rencontrés et leur a fait quelques petites promesses, à mon avis insuffisantes.

Les compétences générales des sages-femmes, définies à l'article L. 4151-1 du code de la santé publique, leur permettent

le Loiret, qui est l'un des départements les plus atteints par la désertification médicale au regard de sa population, compte aujourd'hui 800 médecins de moins que l'Indre-et-Loire, où est implanté le CHU, pour 70 000 habitants de plus. plus. Personne ne comprend les raisons pour lesquelles on ne pourrait pas créer un centre hospitalier universitaire à Orléans, d'autant que les chiffres que nous connaissons montrent que, sur 1 023 médecins en fin d'études, plus de 80 % s'installent à proximité du CHU dans lequel ils ont suivi leur formation.

La mise en place d'un CHU dans un département n'est pas obligatoire et n'est pas non plus obligatoirement synonyme de qualité supplémentaire dans les soins qui peuvent être dispensés par les professionnels hospitaliers qui sont dans les hôpitaux par ailleurs. Il y a quelque temps, la commission

dans le cadre de la mission « CHU de demain ». Si je n'ai pas de réponse défavorable ou favorable à émettre sur un sujet aussi important que celui-là, je pense que

prévalu à la création des CHU. Les ordonnances Debré précisaient que, dans les villes sièges de facultés de médecine, de facultés mixtes de médecine et de pharmacie, les facultés et les centres hospitaliers devaient organiser conjointement l'ensemble de leurs services en en centres de soins d'enseignement et de recherche. Ces centres ont pris le nom de centre hospitalier universitaire. C'est en fait la présence d'une faculté de médecine qui détermine la reconnaissance d'un CHU, et c'est à ce titre que certains chefs-lieux de région ne sont pas siège de CHU à ce jour. Le Gouvernement ne souhaite pas revenir sur cette logique qui fonde la spécificité des CHU, lieu de réunion du soin, de la recherche et de l'enseignement. Il préfère suivre les recommandations de la Cour des comptes et organiser des réseaux entre hôpitaux.

la fin de la Paces, le fait que l'entrée dans les études de médecine puisse se faire à partir de formations universitaires qui ne sont pas des UFR de médecine -diversifieront l'origine des étudiants

avec cet article, qui donne toute latitude au Gouvernement pour redessiner la carte des soins en France, en lui permettant notamment de modifier à sa guise les régimes d'autorisations des activités de soins. L'enjeu de cette réforme est loin d'être purement technique. De son contenu va dépendre en partie la réussite ou l'échec de la mise en place d'une offre de soins hospitalière véritablement territorialisée et graduée, propre à garantir à l'ensemble de la population un égal accès à des soins de qualité délivrés dans des conditions de sécurité optimales. Un encadrement juridique plus strict des conditions d'implantation et de fonctionnement de certaines activités de soins comme la chirurgie pourrait avoir des conséquences sur la capacité de certains hôpitaux à continuer de proposer certaines spécialités, compte compte tenu des contraintes auxquelles ces établissements font face. Si le renforcement de la qualité et de la sécurité des soins est une nécessité incontestable, il doit s'accompagner d'outils de coopération et de mutualisation qui permettront aux établissements les moins bien dotés de s'inscrire dans une filière de soins et de bénéficier des moyens d'assurer une offre hospitalière de premier niveau répondant aux nouvelles conditions techniques techniques de fonctionnement. La création d'une équipe médicale territoriale, qui permettrait notamment de mutualiser les ressources médicales et d'assurer une prise en charge coordonnée à l'échelle de plusieurs établissements, constitue à cet égard une piste intéressante. D'autres pistes pourraient également être explorées, telle la suppression de l'obligation, pour les groupements de coopération sanitaire exploitants, d'exploiter les autorisations sur un site unique, ou encore la création d'une autorisation de projet, à l'image de ce qui existe déjà pour les plateaux mutualisés d'imagerie médicale. En tout état de cause, dans un contexte de grande inégalité territoriale, nous ne pouvons

infrastructures d'accueil et de soins. Cette logique est déjà à l'oeuvre s'agissant des maternités. Les arguments relatifs à la pertinence des soins et à la sécurité sanitaire sont avancés en permanence pour justifier des fermetures,

l'article 9 entraînera la réduction globale de l'offre publique de soins et fragilisera l'égal accès aux soins pour tous. Nous demandons donc la suppression de cet article

évidemment, le recours aux ordonnances sur un sujet aussi important. Les autorisations de soins représentent un fort enjeu pour les territoires. Ce regret étant exprimé, on peut constater

travaillé de manière assumée en coconstruction avec l'ensemble des acteurs. Une partie des travaux entrepris dans le cadre de cette réforme s'achèvera dès cet été, l'autre partie devant être terminée pour la fin de l'année.

Nombre de pays se sont emparés de ces outils pour améliorer la qualité de leurs soins. Nous devons faire évoluer ces critères, comme tous les pays du monde qui travaillent sur les critères de qualité des soins. Telles sont les raisons pour lesquelles je suis défavorable à ces deux amendements. Je mets

Selon le principe de non-affectation des recettes aux dépenses, elles peuvent donc être « fondues » afin de financer toutes sortes d'activités et de dépenses des établissements, et donc pas uniquement celles auxquelles elles sont censées être dévolues. Compte tenu des pressions qui pèsent sur l'hôpital, que nous connaissons tous, la prise en charge psychiatrique en pâtit lourdement. Sans compromettre le statut sanitaire de la prise en charge psychiatrique ni sa nécessaire articulation avec les champs MCO et SSR, un compartimentage du compte de résultat principal en trois volets- MCO, psychiatrie, SSR -garantirait aux autorités de tutelle des établissements de santé la bonne affectation des moyens dans les établissements multiactivités. Une telle mesure, peu complexe à mettre en oeuvre dans sa déclinaison opérationnelle, apparaît d'autant plus opportune qu'elle permettrait de conforter les rapprochements entre établissements dans des GHT structures qui semblent être les plus pertinentes pour favoriser l'articulation et l'adéquation entre les parcours de vie et de soins des personnes. Si nous voulons sanctuariser les budgets de la psychiatrie, nous devons d'abord les identifier. Quel

La mesure proposée est technique. De manière plus générale, des ressources nouvelles pour la psychiatrie sont parallèlement attendues dans le prolongement de la feuille de route

considérablement la situation, alors que je suis en train de modifier complètement le mode de financement des activités de MCO, de psychiatrie et de SSR dans le cadre de la réforme de la tarification. J'émets donc un avis défavorable, même si je comprends l'objectif.

du système de santé de 2016, afin de consolider la dynamique de coopération et d'intégration dans la région. Sa mise en oeuvre améliorera structurellement l'offre de soins dans notre pays en renforçant la coordination entre les acteurs de santé. Il s'agit par par exemple d'éviter les doublons, de mieux identifier les compétences sur le territoire concerné, afin de présenter une offre du meilleur niveau en termes de gestion des ressources humaines médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques.

nous l'avons constaté lors des auditions que notre groupe a organisées : le groupement hospitalier de territoire fait peur aux hôpitaux de proximité. Il faudra donc veiller à avoir de l'ambition pour ces hôpitaux et à ne pas réorganiser les services sans étudier les perspectives de rayonnement des GHT à travers les hôpitaux de proximité.

l'élaboration d'un projet médical consensuel et du respect des demandes des patients et des territoires, ainsi que des conditions de travail des personnels hospitaliers. Nous sommes bien sûr favorables aux démarches de mutualisation, de coopération et de complémentarité, mais les difficultés apparaissent lors de leur mise en oeuvre. L'ambition

garantie ; du rôle des commissions médicales d'établissement en matière de qualité et de sécurité des soins, à l'aune notamment de la création des commissions médicales de groupement ; de l'association des équipes médicales aux projets et à la gestion territoriale- gestion territoriale- à cet égard, comment demander aux personnels de s'investir dans des projets de transformation importants si aucune réponse n'est apportée à leurs problèmes de court terme ? - ; enfin, la situation financière des hôpitaux,

D'après la commission d'enquête de 2018 sur l'égal accès aux soins, la mise en place des GHT par la loi Santé de 2016 a conduit à concentrer l'activité hospitalière dans les grosses structures et à fermer les hôpitaux de proximité. Les GHT sont un outil de gestion des pénuries et de mutualisation des services. Nous sommes pour la coopération, la complémentarité. Cependant, la a entraîné des fermetures de lits, des suppressions de postes, et a fortement détérioré les conditions de travail des personnels hospitaliers et la qualité des soins. De plus,

D'ailleurs, le paragraphe III de cet article habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour permettre aux GHT d'« approfondir l'intégration de leurs instances représentatives ou consultatives » c'est l'application des ordonnances de la loi Travail à la fonction publique hospitalière par la fusion des instances du personnel ! Pour l'ensemble de ces raisons, nous demandons la suppression de cet article. Quel

fait par vous-mêmes et par de nombreux acteurs hospitaliers est que beaucoup d'énergie a été consacrée à améliorer les fonctions de support et l'organisation administrative. Par conséquent, toujours dans l'optique de remettre le projet médical

parfois un siphonnage de leurs ressources par l'établissement support, à rebours de l'objectif initial des GHT. J'entends bien les arguments avancés par le Gouvernement, mais je souhaite que nous restions attentifs à bien associer les établissements à cet acte II des GHT.

à la CME. La politique médicale de qualité et de sécurité des soins doit être élaborée par la commission médicale du groupement avec le concours des établissements. Les Les arguments de Mme la ministre semblent pertinents, mais il faut que chaque établissement avance à son rythme et sans contrainte. La réussite des GHT entraînera des adhésions, mais peut-être seulement à moyen terme. Quel

En effet, les psychologues ne sont pas définis comme appartenant à une profession médicale, représentée par la commission médicale d'établissement, ou à une profession paramédicale, représentée par la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-technique. Cet amendement vise à permettre aux psychologues d'être associés à la composition des commissions médicales de GHT, compte tenu du fait qu'ils ne sont représentés par aucune autre instance.

Toutefois, nous avons tenu à préciser le lien entre la commission médicale de groupement instituée par le texte et les commissions médicales d'établissement, pour faire en sorte que la

mais aux équipes hospitalières, d'élaborer ensemble un projet médical qui sera effectivement partagé. Quel est l'avis de la commission ? Le code

Cet amendement a pour objet d'associer les universités aux activités hospitalo-universitaires prévues dans le cadre de l'association entre le groupement hospitalier de territoire et le centre hospitalier universitaire. Il prévoit également d'associer les universités dans le cadre de la coordination des instituts et des écoles de formation paramédicale du groupement, en lien avec l'« universitarisation » des formations paramédicales et les plans de formation continue et de développement professionnel continu des personnels des établissements. des activités hospitalo-universitaires. Le présent amendement apporte une précision qui paraît utile à la commission, en vue d'associer dans ce cadre les universités du territoire aux activités qui les concernent. La commission souhaiterait toutefois connaître l'avis du Gouvernement.

Les questions liées à l'organisation de l'offre de soins dans les territoires doivent être traitées en concertation avec les élus locaux. Aujourd'hui, ils sont associés aux décisions leur participation au comité territorial des élus locaux. le rôle et l'influence de ce comité restent limités. Toute décision concernant l'organisation hospitalière a un impact important et direct sur la médecine de ville. Elle peut également avoir des conséquences pour le bassin de vie en termes d'emplois et de transports. La qualité des soins proposés à l'hôpital doit demeurer le premier critère de maintien, de déplacement ou de suppression d'un service. Cependant, il est également indispensable de prendre en compte l'ensemble des aspects que je Or, ce sont les élus locaux, notamment les maires, qui sont les plus fins connaisseurs de la situation et des besoins du territoire. En conséquence, il semble indispensable de leur réserver deux places au sein du comité stratégique du GHT.

Les questions liées à l'organisation de l'offre de soins dans les territoires peuvent-elles se traiter sans les élus locaux ? Ces élus sont aujourd'hui cantonnés au sein du comité territorial des élus locaux, instance consultative dont le rôle et l'influence sont limités. La qualité des soins La qualité des soins proposés à l'hôpital doit bien entendu demeurer le premier critère de maintien, de déplacement ou de suppression d'un service. Toutefois, toute décision concernant l'organisation hospitalière a des impacts forts et directs sur le maintien et l'installation des médecins en ville, des pharmaciens, des infirmières et, plus généralement, des personnels de santé. Elle a aussi, bien sûr, des conséquences très fortes en termes d'emploi et de transports, pour ne pas dire d'attractivité. Or ce sont les élus locaux, notamment les maires, qui sont souvent le mieux placés

conduirait à ajouter deux représentants des élus à la composition du comité stratégique du GHT, alors qu'il existe par ailleurs un comité territorial des élus locaux.

a pour objet de compléter les prérogatives du comité territorial des élus locaux afin de l'associer plus étroitement à l'élaboration de la stratégie des GHT. Pour ce faire, le comité territorial des élus locaux pourrait donner un avis sur le projet médical partagé, le projet de soins partagé et les conventions de partenariat et d'association entre le GHT et les autres établissements du territoire.

les prérogatives du comité territorial des élus locaux. Cela va dans le sens d'une meilleure association des élus à la politique hospitalière sur le territoire. La commission

La situation catastrophique actuelle, avec un personnel hospitalier en grande souffrance, subissant de plein fouet la réduction drastique des dépenses de santé et les fermetures d'hôpitaux de proximité, atteste de l'échec des politiques poursuivies ces dernières années. Votre volonté, madame la ministre, de transférer davantage de compétences des établissements de santé vers les GHT montre que vous n'entendez toujours pas pas le cri d'alarme des soignants, qui vous demandent de mettre un terme à cette politique de fermeture d'établissements et de services et de leur redonner les moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice de leurs missions. Par ailleurs, vous décidez de renforcer l'intégration des établissements de santé au sein des GHT, alors même que nous ne disposons toujours d'aucun bilan, depuis leur création en 2016 soit habilité à légiférer par ordonnances sur un point essentiel de cette réforme. Notre groupe ne peut qu'exprimer une profonde inquiétude quant aux orientations politiques et à la méthode choisies par le Gouvernement. L'amendement

trois ans après la réforme, nombreux sont les acteurs hospitaliers à déplorer que les énergies aient pu être majoritairement consacrées à l'optimisation de fonctions de support ou à la gestion administrative. L'ambition générale qui sous-tend l'article 10 est donc de déplacer le centre de gravité des GHT pour priorité aux organisations médicale et soignante, en réponse aux attentes exprimées par les professionnels hospitaliers et les patients. L'une des conditions à remplir est de placer, parmi les compétences obligatoirement mutualisées, la gestion des ressources humaines médicales, pharmaceutiques, odontologiques et maïeutiques. Cela m'apparaît comme une avancée capitale, pour trois raisons. D'abord, il n'y aura plus de pratiques concurrentielles en la matière. Actuellement, en raison de la situation tendue de la démographie médicale, des établissements publics qui partagent pourtant la même stratégie médicale se font concurrence pour le recrutement de médecins, en faisant de la surenchère sur les rémunérations.

Enfin, cela constituera un avantage pour les personnels. L'échelle du GHT offrira davantage de visibilité et d'opportunités en matière de déroulement de carrière. Ces gains en matière Ces gains en matière de coopération, de coordination et d'attractivité me paraissent très importants à préserver. Le modèle cible et l'articulation des compétences en la matière entre « établissements parties » et « établissements supports » sont actuellement en discussion dans le cadre de groupes de travail réunissant les parties prenantes, et je me dois de souligner qu'aucun des qu'aucun des participants- organisations syndicales, conférences ou fédérations hospitalières -n'appelle, à ce stade, à un retour en arrière le rétablissement d'une simple faculté en la matière, comme le prévoit le texte adopté par la commission.

Cela permet d'accompagner les groupements qui souhaitent approfondir leur intégration, sans imposer cette évolution à tous. Dans ces conditions, il semble à la commission que les inquiétudes soulevées par les auteurs de l'amendement n° 321 sont levées,

Ces derniers s'inquiètent d'une perte d'autonomie évidente et des conséquences de la concentration annoncée des moyens dans les hôpitaux supports des GHT. Or, certains établissements parties à un groupement assurent la gestion d'un équipement lourd et/ou l'exercice d'une activité avec une prééminence certaine par rapport à l'établissement support. Ces établissements peuvent décider de la constitution d'un pôle interétablissements géré par l'établissement support, selon l'article L. 6132-3 du code de la santé publique. Cependant, dans la mesure où les établissements sont tous différents et ont des spécialités bien définies, l'efficacité réclame d'orienter la concentration des moyens par pôle vers les centres d'excellence. C'est pourquoi l'objet du présent amendement est de permettre, par voie d'avenant, avec l'accord exprès de l'établissement support, de gérer par délégation un pôle interétablissements afin de recentrer des moyens sur l'établissement qui a depuis longtemps développé une expertise dans le domaine considéré. Quel est l'avis de la commission de la commission ? Cette proposition pourrait constituer un levier de valorisation des établissements parties à un GHT, qui ont parfois le sentiment d'une captation du pouvoir par l'établissement support.

à Mme la ministre. L'objet de cet amendement est de rétablir le droit d'option, au sein du GHT, pour la mutualisation de la stratégie d'investissement. L'article 10 vise à renforcer la dynamique de coopération et d'intégration au sein des GHT, tout en tenant compte de leurs différences de situations et de niveaux de développement. La mesure prévoit notamment de créer un droit d'option pour les GHT volontaires les plus matures, leur permettant d'aller plus loin sur certains sujets. Nous mettons ainsi fin, sauf pour les sujets médicaux, à la logique précédente, qui voulait que tous les GHT avancent au même rythme. l'exercice de ce droit d'option, la commission des affaires sociales a supprimé la possibilité de présenter un programme d'investissement et un plan global de financement pluriannuel unique, et donc de mener en commun, entre les différents sites du GHT, Or maintenir cette possibilité, qui par définition n'est pas une obligation, me paraît essentiel. Il s'agit en effet de permettre aux établissements membres d'un groupement, groupement, lorsqu'ils sont volontaires, de présenter dans un document unique leur stratégie financière et d'investissement pluriannuelle. Cela permettra d'assurer la cohérence des investissements de l'ensemble des hôpitaux membres avec le projet médical partagé du groupement. Je suis attachée au principe du volontariat sur ce sujet, car il faut permettre une application souple et adaptée aux réalités et au niveau de maturité de chacun des GHT.

le principe d'une « banque des investissements », qui permettrait de sortir cette enveloppe de l'Ondam. Étant pris sur les tarifs, les investissements structurels ou courants sont souvent une variable d'ajustement, ce qui obère l'avenir des hôpitaux.

fusionner les commissions médicales d'établissement au sein d'une supra-commission médicale de groupement est contraire à une démocratie sanitaire de proximité telle que nous la défendons. Cela vaut aussi pour les directoires, qui auront également la possibilité de fusionner,

Quand on sait la souffrance au travail qui existe dans les établissements de santé, particulièrement dans les hôpitaux publics, il paraît aberrant de fusionner les seules instances où les problèmes de sécurité et de conditions de travail sont abordés.

les Ehpad sont réticents à intégrer une structure perçue à juste titre comme dominée par l'hôpital. De plus, la mutualisation des fonctions de support liée à l'intégration au GHT en tant qu'établissement partie peut les contraindre à renoncer à travailler avec le secteur économique local.

il est essentiel que la réflexion des GHT sur les filières gériatriques soit partagée avec les Ehpad publics du territoire. C'est pourquoi cet amendement prévoit d'associer les Ehpad publics à l'élaboration du projet médical partagé du GHT, sans qu'ils en soient nécessairement parties.

L'amendement présenté par M. Bonne fait suite au rapport sur les Ehpad qu'il a présenté à la commission des affaires sociales et vise à permettre à ces établissements d'être associés au projet médical partagé du GHT, comme le sont les établissements de psychiatrie.

Il est impossible de continuer dans ces conditions, madame la ministre ! Cette tendance est très fortement marquée par un renforcement de la demande sociale dans les hôpitaux, une part non négligeable des patients accueillis étant en très grande précarité. Les soignants accueillent aux urgences une fraction importante de la population en situation de détresse sociale, ce qui nécessite une prise en charge spécifique.

que physique, peinent à faire reconnaître la spécificité de leur travail. La gestion de la violence, la polyvalence de l'exercice, le manque de lits d'aval, l'augmentation de l'activité sont autant d'éléments qui montrent la difficulté de leur activité. Je rappelle d'ailleurs que la circulaire du 22 juillet 1997 exclut

en tension, un plan de modernisation des urgences, qui sera engagé par les ARS, des financements en cas de situation exceptionnelle de tension, une homogénéisation de la prime

égard au pouvoir grandissant des GHT sur l'offre de soins dans les territoires, il nous semble indispensable d'attribuer aux élus locaux un rôle participatif dans la prise de décisions par ces groupements. Aujourd'hui, leurs représentants qui siègent au sein du comité territorial des élus locaux n'ont qu'une voix consultative ; ils ne prennent donc pas part aux décisions de manière effective. les élus ont une connaissance de la situation sanitaire et sociale de leur territoire qui mérite d'être reconnue et prise en compte dans les décisions des GHT. C'est vers eux que les citoyens se tournent en premier lieu lorsqu'une maternité, un service ou un hôpital de proximité ferme ses portes. Ce sont eux aussi qui constatent le désarroi des personnels de santé, qui ne sont plus à même d'exercer convenablement et dignement leur mission de service public. Ce sont également les élus locaux qui se démènent pour trouver des solutions et des financements afin de répondre à l'urgence sanitaire. Aussi les élus ont-ils toute leur place au sein des conseils de surveillance des GHT.

sociales du Sénat, donne compétence au conseil de surveillance de l'hôpital pour délibérer sur les orientations stratégiques et financières pluriannuelles de l'établissement. Cette disposition me semble remettre en cause les équilibres qui régissent la gouvernance des hôpitaux publics depuis plusieurs années et garantissent leur bon fonctionnement. La loi HPST de 2009 a transformé les conseils d'administration des établissements publics en conseils de surveillance, repositionnant ainsi le rôle de cette instance. La responsabilité de la gestion financière de l'établissement et de la politique d'investissement a été clairement confiée au directeur dans le cadre du directoire. Parallèlement, le conseil de surveillance dispose de prérogatives importantes : il se prononce sur la stratégie et, à ce titre, délibère sur le projet d'établissement. Le code de la santé publique prévoit d'ores et déjà que le conseil de surveillance est informé de l'EPRD, l'état des prévisions de recettes et de dépenses, et du programme d'investissement et qu'il délibère sur les résultats financiers dans le cadre de son rôle de contrôle Le conseil de surveillance dispose également d'un pouvoir d'information générale. Dans ce cadre, il ne me semble pas opportun de lui octroyer un pouvoir de délibération sur les champs propres du directoire, ce qui serait de nature à remettre en cause les équilibres entre les instances des établissements de santé.

la disposition insérée dans le projet de loi par votre commission et devenue l'article 10 , qui prévoit que le directeur communique à la présidence du conseil de surveillance les documents stratégiques et financiers préparatoires et décisionnels nécessaires à l'accomplissement des missions du conseil. Nous devons tous oeuvrer pour que le conseil de surveillance soit respecté dans l'exercice de ses compétences. Quel

mis en oeuvre par l'établissement avec d'autres organismes ayant une activité dans le domaine de la santé, notamment des établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés. Cette proposition est en accord avec les nouveaux objectifs du plan Santé 2022 visant à renforcer la coordination territoriale

Sénat, qui écrivait à l'époque, au sujet de l'article 5 du projet de loi : « On peut douter que, telles que les définit le projet de loi, les compétences du conseil de surveillance lui permettent, de façon satisfaisante, d'influencer la stratégie de l'établissement ou de contrôler sa gestion. de cet amendement, il est proposé de redonner du pouvoir aux élus, qui doivent être en mesure de délibérer sur les décisions qui engagent l'avenir et l'organisation de l'établissement. Quel est l'avis de la commission

les matières suivantes : la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, les acquisitions et aliénations de biens immobiliers, la participation à un GHT, le règlement intérieur de l'établissement. Le conseil de surveillance dispose d'ores et déjà d'un pouvoir de délibération sur les enjeux hautement stratégiques. Je pense par exemple aux délibérations sur le projet d'établissement, sur le projet de fusion ou sur le compte financier. En parallèle, il dispose de prérogatives importantes en matière de suivi et de contrôle. À tout moment, le conseil de surveillance peut opérer des vérifications et des contrôles qu'il juge opportuns. Il peut se faire communiquer des documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En outre, je souhaite rappeler que l'article 10 du projet de loi adopté par votre commission des affaires sociales complète déjà les compétences du conseil de surveillance en prévoyant que « le directeur communique à la présidence du conseil de surveillance les documents stratégiques et financiers préparatoires et décisionnels nécessaires à l'accomplissement des missions du conseil Plus fondamentalement, la loi HPST avait établi des équilibres. Aujourd'hui, il y a des responsabilités partagées. Le directeur, en concertation avec le directoire, s'occupe de la gestion financière, du règlement intérieur, la commission médicale d'établissement de la politique d'amélioration de la qualité des soins. À ce titre, le conseil de surveillance émet des avis sur certaines de ces compétences, et non pas une délibération. Dans ce cadre, il ne me semble pas opportun de lui octroyer un pouvoir de délibération élargi, qui remettrait en cause tous les équilibres entre les instances.

de prendre pleinement le virage du numérique. À cet égard, je tiens à saluer votre engagement et votre détermination, madame la ministre : la feuille de route que vous avez tracée, à la fin du mois d'avril, pour accompagner la transformation numérique de notre système de santé témoigne d'une solide ambition. Elle permettra d'engager l'ensemble des acteurs du secteur, professionnels, établissements, assurance maladie et éditeurs de logiciels, dans une nouvelle dynamique. Je souhaite d'emblée indiquer que, à mon sens, l'article 11, portant sur la réforme du système national des données de santé, le SNDS, et sur la création d'une plateforme des données de santé, la PDS, ne présente pas les risques que certains de nos collègues députés ont cru identifier. D'abord, il élargit le périmètre des données versées au SNDS, ce qui, au vu des enjeux de santé publique, ne peut qu'emporter notre adhésion. Nous avons, à ce titre, contribué en commission à y ajouter le GIR comme donnée de santé essentielle. 11 prévoit certes la possibilité d'intégrer des personnes de droit privé au comité éthique de la nouvelle plateforme des données de santé, qui examinera le caractère d'intérêt public des demandes d'accès. Néanmoins, l'arsenal législatif de la loi Informatique et libertés, auquel le texte ne manque pas de se référer, reste parfaitement opérant, et les garanties qu'il apporte, renforcées par l'Assemblée nationale,

de la gestion du SNDS, qui passe de la CNAM gestionnaire unique à plusieurs responsables de traitement désignés par décret, pose la question du transfert de la compétence jusqu'ici exercée par la seule CNAM. D'autre part, bien qu'elle n'expose pas les données de santé à des risques d'exploitation, je m'interroge sur la suppression de la « finalité d'étude, de recherche et d'évaluation », qui semble ouvrir la voie à d'autres formes de traitement, dont on identifie encore mal la portée. Cela étant, l'article 11 me semble aller

au GIP qui sera financé par un budget annuel de 40 millions d'euros, abondé pour moitié par l'État, à hauteur de 80 millions d'euros sur quatre ans. LeHealth Data Hub,projet de plateforme publique des données de santé, remplacera l'INDS et fonctionnera comme un et fonctionnera comme un guichet unique, sécurisé, pour les centres de recherche, les hôpitaux, les start-up, les laboratoires. Il rassemblera des données médico-administratives, issues notamment de l'assurance maladie, carte Vitale, mais aussi des données cliniques venant d'hôpitaux ou de centres de radiologie. D'autres systèmes de données de santé publics pourront également s'adosser au Health Data Hub. En conséquence, nous allons créer un écosystème qui modernisera l'exploitation des données de santé et fera de la France un leader dans ce domaine. Il élève notre pays au rang des nations avancées en matière de recherche médicale et de numérisation de la santé. Se pose la question de la confidentialité des données, que j'ai déjà évoquée, et celle de l'optimisation des données pour des territoires, comme ceux de l'outre-mer, sont exposées à des maladies tropicales et exclusives. Je fais ici référence aux maladies véhiculées par les moustiques, telles que le zika, la dengue ou le chikungunya, qui ont fortement touché La Réunion et les Antilles françaises. À ce sujet, je tiens d'ailleurs à saluer l'équipe de chercheurs de l'Institut Pasteur à Paris, qui, en collaboration avec l'Institut Pasteur de Guadeloupe, le centre hospitalier universitaire de Guadeloupe, le centre hospitalier universitaire de Martinique, Martinique, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, l'Inserm et le CNRS, a mené une vaste étude d'observation de la population lors de l'épidémie de 2016 aux Antilles françaises.

L'article 11 du projet de loi vise à démultiplier les usages des données de santé en mobilisant les techniques à l'état de l'art de l'intelligence artificielle, tout en préservant un haut niveau de protection de la vie privée. La France pourra ainsi devenir un leader mondial dans ce domaine et, surtout, faire bénéficier les Français des avancées de la médecine rendues possibles grâce à l'intelligence artificielle. Pour cela,

aux données de médecine scolaire, transforme profondément ce système. Ces données ne seront plus rassemblées dans une base unique. Certaines seront appariées au SNDS historique de manière automatisée, et d'autres ne le seront que de façon ponctuelle, pour répondre aux besoins de projets précis. Cette configuration permet d'allier l'agilité et la sécurité nécessaires à nos ambitions. Elle n'est toutefois pas compatible avec l'existence d'un responsable de traitement unique, seul chargé de mettre à disposition les données du SNDS ainsi élargi. La CNAM conservera donc ses compétences sur le SNDS historique et le PDS, comme ses missions le prévoient. Elle sera un acteur majeur pour l'exploitation des nouvelles données du SNDSou pour les utilisations les plus innovantes nécessitant des capacités de calcul renforcées, par exemple, ou le recours à des technologies de pointe. De plus, ce projet élargit les possibilités d'accès aux données du SNDS à l'ensemble des traitements d'intérêt public. L'exigence d'une finalité précise de recherche, d'étude ou d'évaluation est supprimée, ce qui, je l'entends, suscite des inquiétudes. Toutefois, cette exigence constitue à l'heure actuelle un frein pour certains travaux, sans apporter de garanties supplémentaires par rapport aux finalités limitées du SNDS, décrites par ailleurs dans la loi. Cette disposition empêche ainsi de constituer des bases de données pérennes entre les données du SNDS et des données sociales ou des données environnementales, ce qui oblige chaque équipe de recherche à créer de telles bases au cas par cas. Au-delà de la perte de ressources liée à l'absence de mutualisation, cette interdiction conduit à la multiplication de sous-bases, et donc à la dissémination de données. Aussi ai-je souhaité supprimer la « finalité d'étude, de recherche ou d'évaluation », mais j'ai ajouté d'autres garanties dans le texte, notamment en supprimant le dispositif de correspondance permettant la réidentification des personnes à partir des données du SNDS.

la protection de la vie privée. Cet équilibre a d'ailleurs été salué par le Conseil d'État, qui a considéré que « le projet de loi ne méconnaît aucune exigence de valeur constitutionnelle ou conventionnelle, dès lors que le SNDS apporte des garanties suffisantes pour l'utilisation des données auxquelles il donne accès ». J'espère avoir ainsi avoir répondu à certaines interrogations.

ses missions. Elle aura notamment pour rôle de réunir, d'organiser et de mettre à disposition les données du système national des données de santé. Ce nouveau dispositif est censé restructurer une base de données de 1,2 milliard de feuilles de soins et d'à peu près 500 millions d'actes médicaux, dispersés entre les hôpitaux, les cliniques et autres laboratoires de biologie médicale. Pour notre part, nous sommes évidemment favorables à ce que ces données soient mises à la disposition de la recherche publique. Notre crainte principale est qu'apparaisse un nouveau marché des données de santé, qui pourrait profiter essentiellement aux grandes multinationales du numérique, moyennant la monétisation de ces données. Nous craignons que cette base de données publique, financée par l'État, soit gratuitement mise à la disposition des géants du numérique, d'autant que nous avons avons appris que Microsoft était déjà candidat pour héberger les données des patients, tout comme Thales et Atos. Atos. Nous craignons aussi qu'une base unique de données de santé fasse l'objet d'attaques de la cybercriminalité. Ainsi, aux États-Unis, plusieurs millions de dossiers de santé ont été piratés entre 2010 et 2017. Les cybercriminels s'intéressent davantage à notre carte Vitale qu'à notre carte bancaire. Quoique ... Toutes les informations concernant la santé peuvent les intéresser

Je vous remercie,

Cette obligation contrevient manifestement à l'esprit de la loi Touraine de janvier 2016, qui entendait circonscrire l'obligation de certification aux personnes morales de droit privé hébergeant pour le compte de tiers, les textes réglementaires d'application allant même jusqu'à définir une relation contractuelle entre l'hébergeur et son client. De même, elle expose potentiellement ces collectivités à des sanctions pénales, alors même que l'hébergement des données de santé à caractère personnel correspond à leur mission de service public. C'est pourquoi il est proposé de les exclure du champ de l'obligation de certification. Quel est l'avis de la commission commission ? Cet amendement apporte une clarification, que la commission a jugée bienvenue, entre le droit issu de la loi Touraine en matière d'hébergement des données de santé et la déclinaison réglementaire qui en a été faite. Il est en effet prévu, au titre de cette loi, que tout hébergeur de données de santé pour le compte de tiers doit recevoir une habilitation préalable. En application stricte, cette disposition devrait donc s'appliquer aux collectivités territoriales, essentiellement les conseils départementaux qui hébergent des données de santé pour le compte de tiers, quand bien même elles en exercent la tutelle administrative et financière : c'est le cas des MDPH pour les conseils départementaux et des CCAS pour les communes. Cette démarche, pouvant coûter jusqu'à 400 000 euros aux collectivités concernées, me semble superflue à deux titres. les dispositions légales qui régissent l'hébergement des données de santé par des personnes morales de droit public sont déjà précisées dans la loi Informatique et libertés. Ensuite, l'intention du législateur à l'origine de cette habilitation était manifestement le champ aux cas où l'hébergement des données de santé était confié à des personnes morales de droit privé. Les dispositions réglementaires qui évoquent explicitement une relation de client à fournisseur sont, à cet égard, incontestables. La commission est donc favorable

de GIR, qui sont relatives au niveau de perte d'autonomie d'une personne âgée. Cet ajout ouvre des perspectives très pertinentes pour les études sur la dépendance. Toutefois, il ne s'agit pas de données de santé par nature. Les intégrer systématiquement au SNDS reviendrait à leur

Les fichiers de l'assurance maladie, alimentés par les cartes Vitale, ne contiennent pas le diagnostic, seulement le nom des médicaments à rembourser. Il est est donc assez compliqué d'en déduire les pathologies soignées. Néanmoins, si ce fichier est insuffisant en lui-même, il peut être croisé avec d'autres informations, comme celles provenant des hôpitaux ou des laboratoires d'analyses ou d'imagerie médicale, et ainsi constituer une source précieuse pour la recherche. Sans le fichier de l'assurance maladie, la future plateforme des données de santé ne sera pas vraiment alimentée. Pour autant, qui est le propriétaire des informations détenues par l'assurance maladie ?

C'est pourquoi exclure l'assurance maladie du pilotage de la plateforme des données de santé, alors même que c'est elle qui assure la mission, essentielle, de collecte des données, nous paraît assez dangereux et déconnecté des réalités. Notre amendement vise à corriger cette erreur.

CPAM. Plus spécifiquement, il convient de bien distinguer la mission, certes essentielle, qu'assurait jusqu'alors la CNAM comme gestionnaire unique des données de santé du SNDS et la mission de l'Institut national des données de santé, auquel se substitue la PDS, qui a pour tâche de se prononcer qui a pour tâche de se prononcer sur l'opportunité d'une demande de traitement de ces données de santé. La CNAM, contrairement à ce qu'affirment les auteurs de l'amendement, n'assure pas la collecte des données de santé ; elle gère l'entrepôt national alimenté par ses divers contributeurs. Ce monopole de gestion est d'ailleurs abrogé par le présent projet de loi. Cette mission, essentiellement gestionnaire, ne confère pas en soi la qualité à l'organe gestionnaire pour se prononcer sur l'opportunité d'une demande de traitement.

et représentative, constituée de l'État, des organismes assurant une représentation des patients et des usagers du système de santé, des producteurs de données de santé- je pense par exemple aux hôpitaux publics ou aux équipes de recherche du CNRS -, des utilisateurs

des données de santé » : l'État, les organismes assurant une représentation des malades et des usagers du système de santé, des producteurs de données de santé et des utilisateurs publics et privés de données de santé, y compris des organismes de recherche en santé. a pour objet de prévoir que les professionnels de santé qui ont successivement été membres de l'Institut des données de santé puis de l'Institut national des données de santé soient membres de la future plateforme des données de santé. La parole

S'il nous semble normal qu'il soit composé de représentants de l'État, des malades et des usagers ou d'utilisateurs publics, l'expression « utilisateurs privés » nous inquiète. Nous vous demandons, madame la ministre, monsieur le rapporteur, de nous apporter quelques précisions sur ce que

Bien que la commission ne juge pas risquée cette refonte d'ampleur, la multiplication des organismes collecteurs ou des entrepôts de données ne nous semble pas de nature à lever les craintes d'une mauvaise utilisation des données,

plus ou moins habituées à manipuler des données sensibles, induisent mécaniquement une augmentation des risques de fuite de données, par inadvertance- un sous-traitant technique peu exigeant - ou à la suite de manoeuvres crapuleuses Trop nombreux sont les acteurs privés, les sociétés d'assurances notamment, qui voient dans l'acquisition et l'utilisation de ces données de santé un marché très lucratif. L'article cité précédemment relève qu'« il se passe rarement plus de quelques jours sans qu'on ne découvre une faille de sécurité sur des logiciels clés ou, plus grave, qu'une fuite de données ne soit révélée Nous vous alertons de nouveau sur le risque de voir ces données mises sur le marché, comme c'est déjà le cas pour d'autres données à caractère privé. Il s'agit de s'assurer que ces données, trop sensibles pour ne pas bénéficier d'une protection supérieure, soient utilisées exclusivement pour un motif d'intérêt public. Mes chers collègues, collègues, la protection des patients et de leurs données personnelles ne fait pas l'objet d'un clivage politique entre nous. Aussi vous proposons-nous de garantir par voie législative ce droit fondamental.

à l'encontre de la position de la commission, selon laquelle il n'est pas nécessaire d'isoler les demandeurs de traitements de données de santé à caractère commercial, étant donné le maintien de l'impératif de conformité à des référentiels et des méthodologies de référence établis par la CNIL, celui d'un critère nécessaire d'intérêt public pour toute demande de traitement, même à but commercial, et l'exclusion, déjà prévue par la loi, de finalités particulières visant à promouvoir des produits de santé ou à exclure des bénéficiaires de certains contrats

en termes de structuration des données de santé, tout en préservant un haut niveau de protection de la vie privée. Quel est l'avis de la commission

dans le nom du comité chargé de formuler un avis sur les études et recherches dans le domaine de la santé lorsque ces recherches n'impliquent pas la personne humaine. En effet, c'est le caractère d'intérêt public qui conditionne l'autorisation de la CNIL pour ces recherches. Ce critère est essentiel pour assurer la conformité des pratiques au RGPD. La mention de l'intérêt public rendrait le nom du comité plus cohérent avec l'objet de ses missions. C'est pourquoi nous proposons de renommer le comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé « comité d'intérêt public et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans domaine de la santé commission ? Mon cher collègue, il ne me paraît pas opportun de supprimer la mention du terme « éthique » pour l'examen des demandes de traitement de données qui n'ont pas trait à la personne humaine. En effet, de nombreuses demandes de traitement adressées au SNDS prennent pour base des questionnaires identifiables remplis par des patients, que les gestionnaires des données de santé recoupent ensuite avec les données pseudonymisées du SNDS. Pour garantir la sécurité de ces extractions particulières, qui ne concernent pas toutes la personne humaine, mais requièrent tout de même l'avis du Comité de protection des personnes, le CPP, il semble important de maintenir l'examen de la portée éthique de ces demandes. La commission demande

pertinents afin d'inciter les professionnels de santé à produire et à fournir ces données, notamment par le biais des registres adéquats, en respectant les normes de standardisation définies par la plateforme. l'avis de la commission ? Cet amendement vise à attribuer une nouvelle mission à la plateforme des données de santé qui se substituera à l'Institut national des données de santé. que la PDS signera avec les syndicats de médecins des conventions nationales encadrant la collecte et la communication par ces derniers de certaines données de santé relatives notamment aux thérapies innovantes. Cette précision a paru à la commission

pour compléter la logique de coordination développée par cette loi. Pour qu'elle atteigne ses objectifs en termes de santé publique, la plateforme doit aussi ouvrir ses données aux fédérations hospitalières, qui jouent un rôle primordial et peuvent se nourrir de ces données pour améliorer leurs procédures.

de tout statut. Il existe actuellement un régime juridique d'exception qui exonère plusieurs acteurs, énumérés par la loi Informatique et libertés, de la conformité aux référentiels établis par la CNIL et du critère d'intérêt public des demandes de traitement pour accéder aux données de santé. Ces acteurs ont tous pour point commun

ouvrirait une brèche importante dans la sécurité du SNDS. Nous ne manquerions alors pas de retomber dans certains scandales passés, à la faveur desquels des données personnelles se trouvaient accessibles et transmissibles sans contrôle. La commission a donc émis un avis défavorable

différents de ceux pour lesquels elles avaient été initialement fournies ou captées. L'analyse porte sur un nombre de données très important, qui n'a généralement pas été fixé à l'avance. Leur croisement permet souvent une identification très précise des personnes et les efforts d'anonymisation d'anonymisation des données initiales peuvent ne plus constituer une garantie suffisante de la protection des droits de la personne. C'est pourquoi nous n'estimons pas opportun de faire une exception au contrôle de la CNIL pour les traitements de données de santé mis en oeuvre par l'État dans le cadre de l'évaluation des politiques publiques de santé ou à des fins statistiques,

Contrairement à ce qui est suggéré, ce n'est pas parce que les traitements mis en oeuvre par l'État échappent au régime d'autorisation décrit par la sous-section 1 de la section 3 de la loi qu'ils échappent à celui qui est décrit par la sous-section 2.

Les modalités de création et de gestion du Health Data Hub, ou plateforme des données de santé, ne sont pas suffisamment encadrées par le projet de loi. Celui-ci fixe un cadre très général devant permettre au Gouvernement d'avancer sur ce dossier selon une démarche d'incrémentation et d'essais/erreurs.

de l'amendement n° 448, l'instauration, à l'article 12, d'un espace numérique de santé fait de l'usager le gestionnaire unique de ses propres données de santé. Il peut en réguler lui-même les accès sur des applications et des objets connectés dont l'interopérabilité et la sécurité seront assurées par un groupement d'intérêt public. Par ailleurs, l'usage de certaines données de santé à des fins strictement commerciales ou de sélection pour l'éligibilité à certains produits d'assurance est déjà prohibé par le code de la santé publique. Enfin, l'amendement contrevient à l'article 11 A du projet de loi, aux termes duquel l'ensemble des droits sur les données de santé réunies au sein du SNDS restent exercés par l'État. Le code de la santé publique exclut tout exercice d'un droit patrimonial en garantissant l'accès gratuit à ces données sous leur forme agrégée et pseudonymisée. La commission est donc défavorable

Ces zones seront accessibles à tous les acteurs innovants, notamment en intelligence artificielle. Un cadre administratif standardisé sera défini par décret. Des investissements en infrastructures numériques capteurs, réseaux, data centers - permettront à l'ensemble des équipements de santé de fournir des données numériques sur leur usage, des mesures cliniques et biologiques ou des statuts de fonctionnement. telle recommandation vise à créer les conditions permettant de tester des innovations en intelligence artificielle, avec des délais de mise en oeuvre le plus réduits possible. La liste des lieux d'expérimentation serait à la disposition de tous les acteurs souhaitant innover.

l'avis du Gouvernement ? Il s'agit de permettre par la loi au ministre chargé de la santé d'instituer des zones d'expérimentation, afin de développer le recours à l'intelligence artificielle en matière de santé. Le dispositif proposé n'explicite aucune dérogation aux règles en vigueur et n'apporte donc pas de simplification au dispositif actuel d'autorisation de traitement des données de santé. Par ailleurs, il est susceptible de créer une confusion avec les dispositifs déjà existants, notamment la création d'entrepôts de données hospitaliers, conformément à la stratégie du Health Data Hub. Enfin, la rédaction de l'amendement étant trop imprécise quant aux finalités de l'expérimentation et à son champ d'application, elle risque d'être frappée d'inconstitutionnalité. Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à cet amendement.

La collecte de ces données par les gestionnaires du SNDS n'entraîne pas de transfert de propriété. Les droits exercés par l'État sur ces données, reconnus par l'article 11 A, restent d'une nature extrapatrimoniale. Par ailleurs, l'alimentation des données du SNDS sera désormais assurée par plusieurs gestionnaires, et non plus par la seule CNAM, cela dans les conditions énoncées par décret en Conseil d'État. L'État entend donc maintenir l'exercice d'un contrôle sur la seule désignation des gestionnaires de données. Enfin, la loi prévoit déjà l'exercice d'un régime d'accès dérogatoire et inconditionnel aux données de santé pour l'État, ce qui s'avère particulièrement nécessaire et souhaitable dans certains cas, notamment

Parmi eux, le français Doctolib revendique le titre de premier opérateur mondial de plateforme en ligne sur le marché de la prise de rendez-vous médicaux, devant l'américain Zocdoc ou l'indien Practo, et très loin devant ses rivaux français, comme Pages Jaunes, KelDoc ou RDVmédicaux. Afin de prévenir l'irruption de logiques marchandes dans le domaine de la santé, il nous incombe de prendre des mesures à protéger patients et professionnels de santé des pratiques prédatrices et déloyales de certains opérateurs de plateforme. Au regard des graves dérives qui ont entaché l'essor de plateformes similaires, dans le secteur hôtelier en particulier, il convient d'anticiper leur développement afin d'apporter des protections aux médecins et aux patients face aux géants du secteur. D'ores et déjà, chez les opérateurs de plateforme en ligne, il a été constaté le recours à des pratiques anticoncurrentielles et déloyales reposant sur un référencement biaisé des professionnels de santé. En effet, en référençant des professionnels non abonnés, les plateformes redirigent la patientèle de ces professionnels vers certains de leurs propres clients.

La plateforme a procédé au référencement du médecin A afin de pouvoir proposer au patient de recourir à un de ses clients. Ce type de référencement s'effectue sur la base de listings d'anciens clients de ces entreprises. Plus grave, il s'appuie parfois sur le registre de l'ordre des médecins. Ces pratiques contreviennent au règlement général sur la protection des données et, plus largement, au droit européen de la concurrence. Elles vont à l'encontre de la règle de désignation d'un médecin traitant. Aussi cet amendement vise-t-il à proscrire tout référencement de professionnels de santé non abonnés ou ayant résilié leur abonnement. En introduisant à cette fin un article nouveau dans le code de la consommation, nous nous assurerons que les professionnels de la santé ne pâtissent pas de l'hégémonie grandissante de certaines plateformes dont les méthodes lèsent également les patients, qui sont bien souvent les premières victimes de ce jeu de dupes.

prévoit déjà que l'autorité administrative compétente puisse procéder à des enquêtes afin d'évaluer les pratiques des opérateurs de plateforme en ligne. Si celles-ci ne respectent pas le RGPD, elles peuvent être sanctionnées. sanctionnées. Au niveau européen, une proposition de règlement promouvant l'équité et la transparence pour les utilisateurs professionnels des services d'intermédiation en ligne prévoit de renforcer les obligations d'équité, de transparence et de prévisibilité des plateformes à l'égard de leurs utilisateurs professionnels de favoriser le recours à des moyens alternatifs de règlement des différends. Adopter des dispositions franco-françaises spécifiques au cas des plateformes de prise de rendez-vous médicaux en ligne

ont mis en lumière une absence de cadrage effectif des initiatives numériques territoriales, conjuguée aux carences des solutions proposées aujourd'hui par les éditeurs en matière d'interopérabilité.

Cette situation est particulièrement préjudiciable à la coordination et à la continuité des soins. La commission souhaite donc amener les éditeurs à se conformer à des exigences minimales en termes d'interopérabilité. À cet effet, elle a posé le principe d'une labellisation des systèmes d'information et a institué plusieurs mécanismes destinés à les inciter à recourir à cette labellisation. Par ailleurs, notre commission ne souhaite pas que la mise en place de l'espace numérique de santé connaisse les mêmes atermoiements que celle du dossier médical partagé. C'est pourquoi elle a tenu à rendre automatique, pour tout usager du système de santé, l'ouverture de l'espace numérique de santé et du dossier médical partagé. À cet égard, sachons tirer les enseignements d'expériences étrangères inspirantes. Le système de santé estonien a connu une révolution numérique dès 2008. Les résultats de cette politique numérique volontariste ont de quoi intimider aujourd'hui, 99 % des patients estoniens disposent d'une carte d'identité de santé électronique et d'un dossier médical partagé ; 99 % des données de santé et des prescriptions produites par les hôpitaux et les professionnels d'Estonie sont numériques ; 100 % des facturations des frais de santé sont désormais réalisées électroniquement une technologie de est utilisée pour préserver l'intégrité et la sécurité des données de santé. Notre pays, encore une fois, accuse un retard navrant, après avoir pourtant eu très tôt une bonne idée, en lançant le dossier médical partagé dès 2004. Nous ne pouvons plus nous permettre le luxe d'hésiter- je sais que vous partagez ce point de vue, madame la ministre. C'est avec cette exigence que la commission a examiné les dispositions du projet de loi relatives au numérique et les amendements qui s'y rapportent.

A. Effectivement, l'interopérabilité des systèmes d'information est primordiale ; elle est d'ailleurs indispensable à l'utilisation fluide des logiciels par les professionnels et à leur coordination autour d'un patient donné. C'est dans cette optique que j'ai lancé, le 25 avril dernier, à l'occasion de la publication de la feuille de route du chantier numérique de mon plan Ma santé 2022, une action visant à renforcer l'interopérabilité des systèmes d'information. Les modifications apportées par cet amendement s'inscrivent dans cette démarche et permettront aux pouvoirs publics de recourir à des leviers financiers et contractuels à fort impact, pragmatiques et adaptés à l'hétérogénéité de l'écosystème. C'est la raison pour laquelle je suis très favorable à l'amendement

afin que l'attribution de fonds publics soit conditionnée à des engagements de mise en conformité des référentiels d'interopérabilité. que les conventions d'objectifs et de gestion de l'assurance maladie comprennent des engagements relatifs à l'utilisation de systèmes d'information attestés conformes, il est nécessaire que l'obligation de conformité stipulée